nous a plongés, a plongé l'ensemble du pays, dans une grande émotion. La séance, ce matin-là, a été suspendue dès l'annonce de cette triste nouvelle.

à cet homme d'État au parcours exceptionnel, qui a profondément marqué la France et les Français. Nous étions nombreux, sénateurs et anciens sénateurs, à assister avant-hier à la cérémonie d'adieu en l'église Saint-Sulpice.

avait de la France une connaissance intime, celle d'un homme qui a gravi tous les échelons des mandats de terrain avant de présider au destin de la Nation. Né de parents corréziens, Jacques Chirac accomplit ses études primaires et secondaires d'abord à Sainte-Féréole, en Corrèze, puis à Versailles et à Paris. Après son bac, rêvant de faire carrière dans la marine marchande, il s'engagea quelques mois comme pilotin sur un cargo charbonnier, mais son père ne le laissa pas persévérer dans cette voie. Il reprit alors ses études : Sciences Po, puis l'université d'Harvard, enfin l'École nationale d'administration. Au cours de son service militaire, il se porta volontaire pour partir vers l'Algérie en guerre. Cette période d'aspirant, puis de sous-lieutenant, le marquera profondément. Il ira jusqu'à dire qu'elle fut peut-être la plus passionnante de son existence. Si Jacques Chirac débuta sa carrière à la Cour des comptes, très vite, il s'engagea dans la vie politique dès 1962, à trente ans, il devint chargé de mission au secrétariat général du Gouvernement, puis au cabinet du Premier ministre, Georges Pompidou, son mentor en politique, auquel il témoigna une fidélité indéfectible. Parallèlement, avec l'énergie et la ténacité qui le caractérisaient, il se lança à la conquête de la Corrèze, se confrontant avec succès au suffrage universel.

personnelles. Ministre de l'agriculture, Jacques Chirac a profondément marqué le monde agricole, dans une relation exceptionnelle nouée au moment où la politique agricole commune se mettait en place.

Jacques Chirac a incarné les valeurs de notre République. La liberté, d'abord, en refusant toute compromission avec les extrêmes et en assumant le passé de notre pays, ses lumières et ses ombres

d'un Paris qu'il a profondément aimé et transformé, comme de la Corrèze à laquelle il était tellement attaché. La fraternité, enfin, dans sa proximité avec les Français, dans sa sensibilité à la souffrance de ceux qui sont empêchés par le handicap ou la maladie-

fut, comme la sécurité routière, un autre grand chantier de son second mandat présidentiel ; il permit des améliorations dans la lutte contre cette terrible maladie. Sur la scène internationale,

il sut aussi assurer l'adaptation des moyens de notre défense aux progrès techniques et à leurs exigences. Il décida ainsi, ce qui n'était pas simple, la professionnalisation de nos armées. Il chercha à promouvoir le multilatéralisme dans les relations internationales. Portant haut la voix de la France, il n'hésita pas à s'opposer aux Américains : le « non » à la guerre en Irak restera dans l'histoire.

Des textes majeurs furent adoptés en la matière en 1975 et 1976, alors qu'il était Premier ministre, et la Charte de l'environnement fut intégrée au bloc de constitutionnalité en 2004, pendant son second mandat présidentiel. Jacques Chirac était aussi un homme de culture, passionné par l'histoire des civilisations africaines et asiatiques, domaine dans lequel il faisait preuve d'une incroyable érudition. Il nous laisse un grand musée. grand musée. Chaleureux, attentif aux autres, simple aussi, il prenait le temps d'écouter et d'avoir un mot pour chacun, puissant ou humble. Il compatissait aux souffrances d'autrui, mais, pudique et discret, n'évoquait jamais les siennes, alors que la vie ne l'avait pas épargné. Sa profonde humanité, sa proximité avec ses concitoyens et son contact charnel avec les Français ont suscité une sympathie qui dépasse toutes les sensibilités, comme en ont témoigné, dimanche dernier, les interminables files d'attente pour se recueillir devant son cercueil, lors de l'hommage populaire aux Invalides. Permettez-moi de rappeler aussi combien Jacques Chirac aimait la France des outre-mer. Il l'aimait passionnément et avec attention. Il avait parfaitement compris que la France n'est vraiment la France qu'avec ses outre-mer.

à sa fille, Claude Chirac, à son petit-fils, Martin, à toute sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je renouvelle, au nom du Sénat, l'expression de la part que nous prenons à leur chagrin.

Monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs,

Beaucoup a été dit, et très bien dit, sur ce sublime guerrier de la politique, sur son incroyable carrière, sans doute unique en son genre, sur ses victoires à la hussarde, sur ses défaites retentissantes, sur ses erreurs- qui n'en commet pas, surtout durant une si longue carrière ? Beaucoup a été dit, et très bien dit, sur ses intuitions politiques profondes sur ses décisions majeures, que le président Chirac a prises parfois soutenu, parfois seul, et dont nous mesurons aujourd'hui la sagesse et la perspicacité. Beaucoup a été dit, et très bien dit, sur sa personnalité attachante et complexe, sur ses habitudes, sur ses goûts, sur ses combats secrets et ses blessures intimes. Nombre de ces récits proviennent de compagnons,

la politique est parfois brutale, et peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'elle devrait être, elle peut être aussi, quand on le veut, l'expression d'un certain panache et le creuset d'amitiés profondes qui dépassent- c'est heureux -les limites des familles politiques, quand il s'agit de défendre une idée, un territoire, l'intérêt de la Nation ou des valeurs communes. Le Sénat, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, est une excellente incarnation de cette opiniâtreté courtoise- ou de cette courtoisie opiniâtre, je ne sais comment dire -de la République, que Jacques Chirac lui aussi

ans. Ainsi, il aura été à la fois un grand élu de la France rurale et le maire d'une des plus puissantes métropoles d'Europe- deux réalités françaises que Jacques Chirac synthétisait

nous sommes nombreux ici à avoir sillonné une ville, un canton, un département dans tous les sens, aucun d'entre nous, probablement, n'a sillonné la France autant que Jacques Chirac. Nous savons qu'un territoire, ce n'est pas un dossier ; que, pour le connaître, il faut l'arpenter physiquement, mètre carré par mètre carré. quand nous arrivons à destination, après quelques kilomètres d'une route cabossée, dans un lieu comme il en existe des milliers en France- des lieux qui en font bien souvent le charme -, je sais que nous sommes nombreux, quelles que soient nos opinions politiques,

au moment où les responsables politiques de l'Hexagone et des outre-mer, avec des chefs d'État du monde entier, se recueillaient en l'église Saint-Sulpice, nos compatriotes et leurs élus rendaient, eux aussi, hommage à Jacques Chirac : des centaines de personnes se sont réunies place de la République à Mamoudzou, à Mayotte, ainsi qu'au jardin de l'État à Saint-Denis de La Réunion ; des minutes de silence ont été observées en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Wallis-et-Futuna les habitants de Nouvelle-Calédonie ont pu exprimer leur émotion dans plusieurs livres d'or. Les unes des quotidiens d'outre-mer sont particulièrement éloquentes, où les mêmes termes reviennent : l'amoureux, l'ami, le grand défenseur.

Un grand nombre de Calédoniens se souviennent que c'est sous l'autorité du même Jacques Chirac que la République a adopté la révision constitutionnelle gelant le corps électoral pour les élections provinciales. Au reste, j'observe que responsables indépendantistes et non indépendantistes ont salué avec une même émotion la mémoire du président défunt. Gardons également en mémoire la décision difficile, car éminemment stratégique, de relancer les essais nucléaires en Polynésie française : une décision qui a provoqué des contestations, parfois violentes,

Il ne l'a jamais été, ce qui ne l'a pas empêché de bien connaître votre assemblée, comme ministre chargé des relations avec le Parlement, puis comme Premier ministre. Dans une courte intervention pour accueillir les membres du bureau du Sénat à l'Élysée, en 1995, Jacques Chirac rappelait ainsi qu'il avait toujours entretenu des relations courtoises avec le Sénat.

Un enracinement profond, une attention particulière aux territoires de la République, un amour de nos terroirs : voilà ce qui a fait de Jacques Chirac l'incarnation de la France et des Français- de nous tous, en somme -, avec ce que cela implique de défauts, de générosité et parfois de génie. Pour paraphraser Malraux, le patriotisme de Jacques Chirac ignorait le chauvinisme. Cet équilibre subtil, exigeant, c'est celui d'une France souveraine, autonome, farouchement indépendante, d'une France fière de son identité, mais capable de s'ouvrir et de parler à tous, avec raison, mesure et sagesse ; de la France du multilatéralisme, du projet européen et de l'amitié franco-allemande,

Dans l'une de ses dernières interventions, en mars 2017, le président Jacques Chirac nous exhortait à refuser l'extrémisme sous toutes ses formes. Douze ans plus tard, nous savons que ces propos n'ont rien perdu de leur acuité ; ils nous placent chacun devant nos responsabilités.

Ils l'aiment comme on aime parfois ceux qui vous ressemblent le plus : avec des intermittences, des impatiences, mais aussi avec une profonde tendresse et une fidélité peu commune, qui résiste à tout. Aux vicissitudes de la vie politique, aux erreurs, aux opinions du moment. Et, surtout, au temps. Monsieur le

de la Seine-Maritime et au-delà. Je remercie vivement les forces de l'ordre, les salariés de l'usine et nos pompiers, car le pire a été évité. Mais, chez les habitants, une angoisse et une colère Les enquêtes judiciaire et administrative doivent rapidement déterminer les responsabilités. Mais, à cette heure, c'est la santé qui prime : à cet égard, des réponses précises et des explications claires sont attendues. Lors de votre visite sur place, monsieur le Premier ministre, vous vous êtes engagé à la transparence, du reste garantie par l'article 7 de la Charte de l'environnement. hier, le préfet a dévoilé des chiffres alarmants : 5 253 tonnes de produits chimiques ont été brûlées et 160 fûts sont toujours entreposés, dans un état délicat. Il faut que les prochaines analyses nous renseignent sur les molécules dégagées qui ont été inhalées, les retombées de suie et leurs conséquences ! Nos familles sont inquiètes. Vous avez reconnu la nécessité d'un suivi médical de long terme, mais il faut aussi un suivi épidémiologique strict de ceux qui sont intervenus sur le sinistre et de toute la population touchée d'une manière ou d'une autre. Si, comme vous le dites, la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique n'est pas envisagée, quelle solution proposez-vous pour indemniser les victimes ? Je remercie Didier Guillaume, qui a reconnu la gravité de la situation et promis des aides aux agriculteurs, éleveurs et maraîchers des 206 communes de Normandie et des Hauts-de-France concernées par la suspension des récoltes et des collectes de lait. Enfin, lorsqu'un événement de cette gravité et de cette ampleur se produit, il faut que l'ensemble des maires soient bien informés. Or ils nous ont dit regretter de n'avoir pas toujours pu jouer leur rôle auprès de la population.

très spectaculaire et grave a été maîtrisé en douze heures, sans victime ni blessé,

Je redis le plus clairement et le plus fermement possible l'engagement absolu du Gouvernement à la transparence totale, complète. Toutes les informations, toutes les données scientifiques qui seront rendues disponibles par les analyses mises en oeuvre seront communiquées au public. Le

car son action était délicate, a reconnu lui-même, lors d'une rencontre avec les maires de la métropole rouennaise, que la qualité de l'information diffusée aux premières heures de l'événement à destination d'un certain nombre de maires n'avait peut-être pas été à la hauteur des aspirations

point. Les consignes de vigilance ont été immédiatement données. Nous avons fait procéder au nettoyage de toutes les écoles avant leur réouverture lundi. Une campagne de surveillance approfondie de l'ensemble des impacts environnementaux sur l'eau, sur l'air, sur les sols avec des prélèvements a commencé dès vendredi. Les résultats sont et seront rendus publics au fur et à mesure de leur délivrance, en fonction des produits qui sont testés et de la difficulté technique de ces analyses, certaines pouvant prendre

un expert de Santé publique France et le chef du service de pneumologie du CHU de Rouen seront associés à ses prises de parole, afin de donner les réponses les plus précises possible aux questions qui ne manqueront pas d'être posées. Hier, en fin d'après-midi, le préfet a rendu publique la liste complète des produits présents dans l'entrepôt qui a brûlé avec les caractéristiques de ces produits et les risques associés. Je veux sur ce point être clair, mesdames, messieurs les sénateurs : depuis la fin de l'année 2017, pour des raisons de sécurité qui n'échapperont à personne, la liste complète des substances autorisées sur les sites classés Seveso n'était plus rendue publique, mais, dans tous les cas, dans tous les cas, cette liste ne dit rien des produits et des quantités qui sont réellement présents sur un site à un moment donné. La liste que nous avons rendue publique hier est précise

c'est que tous les prélèvements d'air dont nous disposons à cette heure, dont les analyses ont été rendues publiques, font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire à l'extérieur du site. Des analyses complémentaires ont été engagées pour vérifier si des fibres d'amiante sont présentes dans l'air, parce que la toiture des bâtiments qui ont brûlé en contenait. Les premiers résultats,

D'autres résultats sur des zones plus éloignées vont suivre dans les prochains jours ; ils seront bien sûr rendus publics. Je n'ignore pas les odeurs incommodantes qui perduraient encore hier.

Les services de l'État travaillent d'ailleurs avec l'entreprise pour résorber les sources d'odeurs. Comme l'a indiqué le préfet hier, les opérations de nettoyage du site sont en cours ; une protection sera installée sur la zone contenant des fûts endommagés pour capter les flux d'air.

La loi Bachelot de 2003, qui a créé cette possibilité, a mis en place un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques. Ce régime, je le dis au Sénat, vise à faciliter le traitement des accidents qui ont eu un très fort impact sur les biens immobiliers et mobiliers en s'appuyant sur le précédent d'AZF à Toulouse en 2001 : des milliers de logements avaient alors été affectés, voire rendus inutilisables.

des riverains et de l'ensemble de ceux qui subissent un préjudice ou un dommage. Je veillerai à ce que rien ne vienne exonérer la responsabilité de l'industriel, car en matière d'installations classées, le régime juridique

qui concerne la transparence, le Gouvernement mettra tout en oeuvre pour dire, pour mesurer et pour faire connaître l'ensemble des causes et des conséquences de cette catastrophe industrielle dont nous souhaitons- nous allons y veiller -qu'elle ne devienne pas une catastrophe sanitaire ou une catastrophe environnementale. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le temps que j'ai pris pour répondre à cette question, mais il me semblait important d'aller jusqu'au bout. La parole est à Mme

pour progresser et faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise pas. La parole

Pour reprendre votre expression, vous souhaitez faire du « cousu main ». Vous avez raison : il existe non plus une seule ruralité, mais plusieurs formes de ruralité, depuis l'hyper-rural jusqu'au périurbain en passant par la montagne. qu'ancien maire d'une commune rurale, Châbons, et d'un bourg-centre, le Grand-Lemps, j'accueille donc ce plan avec beaucoup d'espoir. Espoir, car de nombreuses mesures annoncées sont attendues depuis longtemps la revitalisation des centralités, avec le soutien aux petits commerces, le développement des lieux de convivialité, notamment l'opération 1 000 cafés dans les villages, ou encore le renforcement de l'accompagnement de la jeunesse de ces territoires, en lui facilitant l'accès aux services dont elle n'a pas toujours connaissance- les cartes de réduction, le permis à un euro, etc. -et d'autres propositions relatives à la culture, à l'accès au numérique ou à notre système de santé. bien, madame la ministre : après le temps des annonces doit venir le temps des actes concrets. Afin de garantir la bonne réalisation des mesures de ce plan d'action, pouvez-vous nous préciser la méthode employée pour définir la carte de géographie prioritaire des ruralités, ainsi que le calendrier de cet agenda ? Quand ces territoires pourront-ils concrètement en ressentir les effets et répondre à des appels à projets ? La parole

Et il faut effectivement passer des annonces aux actes concrets pour améliorer la vie quotidienne des habitants de nos campagnes. Pour y parvenir, vous l'avez rappelé, nous avons donné suite à un grand nombre de propositions de la mission agenda rural, dont je tiens à à saluer la qualité du travail. La mission avait notamment recommandé d'élaborer une géographie prioritaire des territoires ruraux. Le Gouvernement a décidé de suivre cette recommandation, car nous pensons qu'il est nécessaire de concentrer nos efforts dans les territoires qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, vous le savez, il existe des zones de revitalisation rurale, les fameuses ZRR, qui sont importantes pour les territoires. Elles couvrent près d'une commune sur deux dans notre pays, et leur effet nécessite d'être évalué. Vous êtes d'ailleurs un certain nombre sur ces travées à partager ce point de vue-je pense en particulier à Bernard Delcros, Frédérique Espagnac et Rémy Pointereau qui viennent de rendre un rapport sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avons pris deux décisions : tout d'abord, prolonger jusqu'à la fin de l'année 2020 le zonage ZRR pour les 4 074 communes qui devaient en sortir en juin prochain ; ensuite, travailler sur une nouvelle géographie prioritaire. Nous avons une année pour le faire, et je le dis dès à présent : cette nouvelle géographie prioritaire sera naturellement définie en lien avec les membres de la mission, mais aussi les associations d'élus, et bien sûr des parlementaires. La méthode du Gouvernement est constante : partir des besoins des territoires et coconstruire les solutions avec ceux qui les représentent.

a formulé 41 recommandations pour répondre à cette problématique. La première conséquence des dérives sectaires dans le domaine de la santé est un nombre important de décès prématurés chaque année ; personne ne peut l'ignorer. Ne nous y trompons pas : ce phénomène touche toute la société et justifie pleinement l'existence de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, créée en 1996 sous une première forme. Son efficacité n'est plus à démontrer. Récemment encore, c'est elle qui a révélé l'affaire des essais cliniques non autorisés sur 350 personnes souffrant des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Ce service, disposant d'un savoir-faire que de nombreux pays nous envient, est considéré comme unique au monde, parce qu'il est à la fois observatoire et régulateur.

auprès du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation ou du bureau central des cultes. Ce rattachement a d'ailleurs déjà été évoqué ou suggéré par la Cour des comptes en 2017. Il semblerait que ce rattachement au titre de la police administrative de la prévention ait été récemment confirmé par le ministère de l'intérieur. Est-ce à penser que la Miviludes perdrait, de fait, ses pouvoirs en matière de police judiciaire ? matière de police judiciaire ? La Miviludes est indispensable dans notre société, touchée à tous les niveaux par les dérives sectaires et les phénomènes d'emprise mentale. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais- et je ne suis pas le seul sur ces travées -connaître vos intentions quant à l'avenir de la Miviludes

d'abord, celle d'analyser le phénomène des dérives sectaires, qui, vous le savez, est mouvant, évolutif-nous l'avons observé au cours de ces vingt dernières années ; ensuite, celle d'assurer la coordination de la politique préventive et répressive de la lutte contre les dérives sectaires ; enfin, la Miviludes joue un rôle extrêmement important en matière de formation des agents publics, et d'une manière générale, de sensibilisation du public sur ce que sont les dérives sectaires.

Troisièmement, et c'est une remarque de bonne administration, de bonne gestion, il est de bonne politique que les politiques publiques soient menées dans les ministères sous l'impulsion et la coordination du Premier ministre

La détermination du Gouvernement à lutter contre le phénomène des dérives sectaires reste pleine et entière. citoyen et écologiste. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, vous avez enfin accepté de publier la liste des produits stockés chez Lubrizol, mais j'imagine et j'espère que les services de l'État en disposaient Alors, pourquoi ne pas avoir fait évaluer dès les premières heures de l'incendie les conséquences sur la santé humaine et des animaux, sur l'air, l'eau, les sols ou les cultures de la combustion de ce cocktail de substances ? Face aux effets sur la santé des populations touchées, quel plan d'action sanitaire, quel suivi épidémiologique comptez-vous concrètement mettre en oeuvre ? Qu'est-il prévu pour les salariés présents sur le site lors de l'incendie, pour les sapeurs-pompiers ou les forces de l'ordre qui sont intervenus, qui ont mis leur vie en jeu et qui ont souvent l'impression, comme nos concitoyens, qu'ils courent de grands risques ? Les élus locaux seront finalement réunis comme nous le demandions. Pouvez-vous nous garantir qu'ils seront désormais consultés et associés à chaque nouvelle étape ? Leur mise à l'écart, l'isolement et même le mépris qu'ils ont ressenti sont inacceptables, mais surtout contre-productifs. Vous vous êtes privés d'acteurs majeurs dans la gestion de la crise. L'usine Lubrizol a bénéficié de ce que vous appelez des « simplifications » de la législation. Il s'agit en réalité d'un détricotage du droit de l'environnement et d'un recul sur les exigences de sûreté, en l'occurrence l'augmentation des stocks sans étude de danger. Allez-vous abandonner vos projets d'alléger encore les obligations d'évaluation environnementale pour les sites

comme le Premier ministre et d'autres collègues, je me suis rendue sur le site. Je mesure donc pleinement à la fois l'émotion et l'inquiétude des populations qui ont été touchées par cette catastrophe industrielle. de vous redire l'engagement du Gouvernement à agir avec la plus grande exigence et dans une transparence totale. C'est dans cet esprit que, dès le début de l'incendie,

déposées. Cette surveillance de l'environnement a été effectuée depuis le départ. Les analyses dont nous disposons aujourd'hui ont fait apparaître qu'il n'y avait pas de

Cette liste a dû être établie à notre demande par l'industriel, parce que, comme vous le savez, les autorisations, qui ne sont au demeurant plus publiques pour les raisons exprimées par le Premier ministre, portent sur la totalité du site. Or ce qui était requis, c'était la liste des produits présents sur la partie incendiée du site. Celle-ci a été diffusée

! La parole est à M. Didier Marie, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, permettez-moi d'associer à mon intervention Nelly Tocqueville, sénatrice de Seine-Maritime, et mes collègues des Hauts-de-France. Il y a six jours, l'agglomération de Rouen a vécu la plus importante catastrophe industrielle connue depuis le drame d'AZF en 2001. L'incendie de l'usine Lubrizol a généré un gigantesque nuage de fumée noire épaisse et nauséabonde, dont les particules ont tapissé jardins, cours d'école, habitations et récoltes, constituant une véritable marée noire terrestre. Le pire a été évité grâce au courage de 240 sapeurs-pompiers et au personnel de l'usine, dont je salue le dévouement. Mais, monsieur le Premier ministre, la gestion de cette crise n'a pas été satisfaisante. Les maires ont été livrés à eux-mêmes : sirènes d'alerte actionnées tardivement, absence d'information dans certaines communes pourtant très proches du sinistre, consignes de confinement confuses, cacophonie totale quant à l'ouverture ou la fermeture des établissements scolaires. Les communications distillées au fil des heures se voulaient rassurantes : elles ont produit l'effet inverse, et la colère a empli le vide d'informations. Comment croire qu'il n'y a pas de danger quand le préfet annonce qu'il n'y a pas de risque de toxicité aiguë, reconnaissant implicitement que les fumées sont bien toxiques ? Comment accepter qu'il n'y ait aucun risque lorsque l'État publie tardivement la liste des produits partis en fumée, et que l'on n'en connaît ni la quantité, ni la résistance à la chaleur, ni la dangerosité ? Comment se sentir en sécurité quand il reste 165 fûts endommagés qui peuvent dégager du sulfure d'hydrogène hautement toxique ? Comment être rassuré lorsque les agriculteurs de 206 communes ne sont toujours pas autorisés à procéder aux récoltes ni à vendre leur lait et leurs produits agricoles ? Monsieur le Premier ministre, pour apaiser la colère et les angoisses, nous vous demandons d'accéder aux demandes suivantes : la transparence- vous y êtes engagé, nous vous en remercions ; la nomination d'un comité d'experts indépendants chargé d'analyser et d'interpréter les résultats des études ; la mise en place d'un suivi médical à court et long terme ; la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique, qui permettrait d'ouvrir droit à indemnisation, même si les biens n'ont pas été détruits ; la réparation rapide des dommages, en ordonnant au préfet d'exercer ses prérogatives de police administrative et d'appliquer le principe du pollueur-payeur, sans attendre l'issue des procédures judiciaires qui prendront des années. Il faut rétablir la confiance et la sérénité en faisant preuve de sérieux et de responsabilité. Ces propositions formulées en association avec une centaine d'élus peuvent y contribuer.

nous les avons. J'ai parfaitement conscience qu'au fur et à mesure que nous diffusons des informations de nouvelles questions se posent. C'est bien naturel, et nous ne nous arrêterons pas à cela, au contraire : toutes les informations qui seront connues seront rendues publiques ; elles susciteront de nouvelles interrogations, de nouvelles interrogations, parfois peut-être de nouvelles angoisses, et nous y répondrons. J'ai parfaitement conscience que la parole et parfois l'expertise publiques sont contestées,

commencer à raconter n'importe quoi ou arrêter de donner les informations pour autant. Nous allons faire exactement ce que je me suis engagé à faire : communiquer au fur et à mesure qu'elles sont disponibles absolument toutes les informations. Pour répondre aux demandes que vous avez formulées,

Cette discussion ne me fait pas peur : elle est nécessaire, elle aura lieu, et nous nous expliquerons. Vous m'interrogez sur la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique. Je comprends bien l'intérêt qu'il pourrait y avoir à reconnaître officiellement qu'une catastrophe a eu lieu. À l'évidence, une catastrophe a eu lieu, mais l'instrument juridique tel qu'il a été conçu par le Parlement en 2003 ne répond manifestement ni

Nous allons donc appliquer toute la loi en la matière, avec la rigueur et avec la totale transparence qui est due à nos concitoyens.

et, peut-être bientôt, du monde. Google détient 90 % du marché des moteurs de recherche. Facebook absorbe les deux tiers des publicités sur internet. Amazon concentre la moitié des ventes en ligne aux États-Unis. En commençant à fixer un cadre et des règles à ces nouveaux empires, la France s'est attiré la fronde des firmes concernées et l'hostilité du président des États-Unis qui nous menace de rétorsion sur les vins français. Hier, Amazon a mis en oeuvre sa menace de reporter sur les vendeurs de sa plateforme la taxe GAFA adoptée le 11 juillet dernier ; 10 000 PME se retrouvent pieds et poings liés, et certaines devront fermer leurs portes. Le 24 octobre prochain, Google entamera un bras de fer contre la nouvelle loi française relative aux droits voisins, qui prévoit une redistribution des revenus du numérique au profit des éditeurs de presse. L'objectif de Google est de forcer les éditeurs à céder tous leurs droits et de faire pression sur les autres gouvernements européens pour une transposition plus favorable de la directive européenne. Monsieur le Premier ministre, le Sherman Act américain de 1890 et les règles européennes contre les abus de position dominante ne sont plus adaptés aux pratiques des Gafam - Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Confisquer les données de la vie privée, racheter les start-up concurrentes, exclure ses rivaux de la publicité en ligne, piller la production des entreprises de presse, ce n'est plus du tout la même chose que capter 90 % du marché du dentifrice. Aujourd'hui, les monopoles des Gafam sont sans doute beaucoup plus préoccupants que ne l'étaient celui de la Standard Oil en 1911 et celui de AT&T en 1982. Des deux côtés de l'Atlantique, de nouvelles lois antitrust sont nécessaires et de plus en plus évoquées. Il est urgent que l'Europe se saisisse de ce dossier. Quelle est la position du gouvernement français à ce sujet ? La parole est à M. le Premier ministre.

La semaine dernière, Google a présenté un nouvel outil de publication pour les éditeurs et les agences de presse. Celui-ci, comme par hasard, a été configuré de telle sorte qu'il n'ouvre pas droit à rémunération, contrairement aux principes posés par la loi du 25 juillet 2019 sur les droits voisins. Ces deux faits, qui ne sont pas sans lien, posent une question juridique, économique et, en vérité, politique extrêmement sérieuse. Pour l'ensemble de nos concitoyens, il n'est pas acceptable qu'un acteur, aussi puissant soit-il- en l'occurrence, ces deux acteurs sont extrêmement puissants -, puisse changer ses règles de publication de manière unilatérale pour contourner une obligation légale.

permettre un juste partage de la valeur produite au bénéfice des plateformes par les contenus et services qu'elles référencent, valeur qui leur procure des revenus qu'elles conservent aujourd'hui en quasi-totalité, voire en totalité. Mesdames, messieurs les sénateurs, en France et en Europe, il existe des entreprises qui innovent et qui créent de la valeur. Il y a aussi des gouvernements qui sont démocratiquement élus. Les lois sont votées par les représentations nationales. Les entreprises doivent mesurer que, en s'y opposant, c'est aux citoyens libres de ces États qu'elles s'opposent. Nous voulons vraiment Nous voulons vraiment croire que la démarche de Google relève de l'erreur d'appréciation, et non de la volonté d'engager une épreuve de force avec la France et l'Europe.

Si nous voulons construire l'espace souverain de droits et de libertés que nous souhaitons bâtir ensemble à l'heure du numérique, alors l'Union européenne, au moins autant que chacun des États qui la composent, doit se saisir du sujet.

membres de la future Commission européenne, et c'est l'un des points qui s'est trouvé au coeur de la discussion entre le Président de la République et la future présidente de la Commission. Ce ne sera pas un combat facile, car nous avons en face de nous des gens déterminés et puissants. Mais ce dont il s'agit, c'est quand même de faire respecter notre souveraineté et notre conception du monde numérique. Ce n'est pas un petit combat ; c'est un combat difficile qu'il nous revient de livrer

Pis, vous aggravez le mal ! Vous remettez en cause plusieurs principes fondamentaux qui constituent, à nos yeux, le coeur de notre système de protection sociale. Vous mettez fin à l'autonomie de la sécurité sociale en ne respectant pas la loi Veil de 1994 et en la privant de près de 3 milliards d'euros avec la mise en oeuvre des mesures d'urgence économiques et sociales en réponse à la crise des gilets jaunes. Par ailleurs, vous mettez fin à son universalité. En matière de politique familiale, alors que la branche famille est excédentaire, vous ne saisissez pas cette opportunité pour relancer politique et redonner confiance aux familles. Bien au contraire, vous persévérez dans la « casse » déjà engagée depuis plusieurs années de notre politique familiale, en prévoyant le quasi-gel des aides aux familles. Enfin, les décisions du Gouvernement en matière de retraite nous laissent pantois quant à sa volonté de ramener l'équilibre du système à court terme. Madame la secrétaire d'État, ma question est la suivante : le Gouvernement entend-il uniquement agir sur le levier de la baisse des pensions d'aujourd'hui et de demain ?

Ces éléments et la révision des perspectives de croissance nous conduisent aujourd'hui à retarder le retour à l'équilibre. Mais notre ambition demeure la même : l'objectif du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux et de désendettement de la sécurité sociale reste entier. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 s'inscrit dans la perspective de la poursuite de l'effort engagé depuis 2018 en matière de maîtrise des dépenses sociales, tout comme pour l'ensemble des dépenses publiques, tout en veillant à préserver et à soutenir nos concitoyens modestes et fragiles.

Milon, pour la réplique. Je voudrais que chacun d'entre nous ait en tête cette déclaration de Simone Veil : « la sécurité sociale, c'est d'abord un immense progrès social et le plus puissant facteur de cohésion sociale qui existe en France ; nous avons le devoir de la préserver pour les générations futures

les pompiers, les personnels des hôpitaux, les enseignants crient eux aussi leur désespoir. Agressions, violences verbales et physiques, menaces, eux aussi sont seuls pour affronter ces tensions quotidiennes.

et détermination aux événements que le Gouvernement ne sait pas maîtriser. Mais la résistance humaine a ses limites Faute de réponse, faute d'une politique sans concession vis-à-vis de la violence, nous assistons à une perte d'autorité sans précédent. Le sentiment d'abandon par la puissance publique domine. Or, monsieur le ministre, un État qui ne protège protège pas ses serviteurs est un navire sans boussole et, donc, en perdition. Quelles sont les mesures immédiates que vous comptez prendre pour protéger les forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction ? Quand vous déciderez-vous à sanctionner ceux qui appellent à la violence et à la mort de tous ces serviteurs qui incarnent pourtant l'autorité de la République ?

dix-huit ans de déficit, la sécurité sociale dégagerait un excédent de 700 millions d'euros en 2019. Nous y sommes

Le projet 2020 intègre-t-il des crédits exceptionnels pour résoudre la crise de l'hôpital ? Avec un Ondam à 2,3 % couplé à 4 milliards d'euros d'économies, ce n'est pas le cas Il y a un an encore, le Gouvernement se préparait à transférer les excédents attendus de la sécurité sociale vers le budget de l'État, fait- « pillage », diront certains -sans précédent.

Ce texte renforce également la prise en compte des nouveaux risques sociaux qui pèsent sur les Français, dont la couverture est l'essence même de la sécurité sociale. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de ces belles mesures que comporte ce projet de loi. Celui-ci prévoit un accompagnement des familles monoparentales, en offrant aux parents séparés un dispositif de sécurisation du versement des pensions alimentaires : plus de 40 millions d'euros seront consacrés à cette mesure dès 2020. Il prévoit aussi la création d'un parcours d'accompagnement après la maladie pour les patients atteints d'un cancer, la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des maladies professionnelles liées aux pesticides,

Nous entendons la demande d'un système social plus juste sans remettre en cause les objectifs du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux. Lors des débats parlementaires, monsieur le sénateur, vous verrez que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 poursuit l'effort important, engagé depuis 2018, de maîtrise des dépenses sociales, comme pour l'ensemble des dépenses publiques, tout en veillant à préserver et à soutenir les citoyens les plus fragiles.

venir de nouveaux coups portés à notre protection sociale ? La sécurité sociale est une assurance solidaire de toute la société. Elle ne saurait en aucun cas se réduire à une chambre de compensation des politiques de l'État ! La parole La parole est à M. Jean-François Husson, pour le groupe Les Républicains. Quatre questions au Gouvernement démontrent la gravité de la situation à la suite de l'incendie de plus de 5 000 tonnes de produits chimiques dans l'usine Lubrizol de Rouen. Il convient de prendre la pleine mesure des conséquences sanitaires et des vives inquiétudes écologiques et économiques qu'expriment les populations et les professionnels intervenus sur le site. Des réponses claires et sans ambiguïté qui relèvent de l'État se sont par trop fait attendre. Une communication brouillonne, inappropriée et inadaptée a donné le sentiment d'une crise très mal gérée par les pouvoirs publics, ce qui ne fait qu'accroître le malaise. Trop de questions restent sans réponse. Aussi, je vous demande, madame la ministre, de faire la lumière sur plusieurs zones d'ombre. Les leçons de l'incident survenu en 2013 ont-elles été tirées et, si tel est le cas, selon quel plan d'action ? Les réglementations Seveso ont-elles été intégralement respectées et, si tel est le cas, sont-elles à la hauteur des défis sanitaires ? Pourquoi avoir attendu cinq longues journées pour publier la liste des produits chimiques présents sur le site de l'usine Lubrizol ?

aux pompiers et aux services qui ont été mobilisés dès le début de l'incendie, qui ont permis de maîtriser ce dernier et d'éviter tout suraccident dans un contexte pourtant très compliqué. Je peux vous assurer que les services de l'État sur le terrain ont également été mobilisés pour réaliser ou faire réaliser par l'exploitant, comme le lui impose la loi, de nombreux prélèvements dans l'air, l'eau, les sols et sur les végétaux.

les services de secours, les services de l'État ne disposaient pas des moyens de faire effectuer des prélèvements et des analyses avec autant de réactivité qu'aujourd'hui. Si nous avons pu disposer de ces informations aussi rapidement, c'est bien parce que nous avons tiré les conséquences de cet incident.

Entretenir le flou par la cacophonie et les déclarations officielles contradictoires n'est pas acceptable et symbolise une crise ingérable face au discrédit de la parole publique.

l'opinion. Enfin, les préoccupations écologiques et environnementales, parce qu'elles sont aujourd'hui entrées dans la conscience des Français, méritent que l'on en partage les défis et les enjeux en toute transparence. Nous avons, l'État au premier chef, un devoir de vérité. Chacun le constatera, il reste beaucoup à faire

civile. Le Premier ministre a rendu un hommage bien légitime aux qualités et à la détermination de nos sapeurs-pompiers, ... Il a bien fait ! ... mais nos sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont à bout de souffle Ces hommes et ces femmes, dont l'engagement au service de nos concitoyens force le respect, sont sur tous les fronts et doivent faire face à une sursollicitation en intervenant parfois, et de plus en plus souvent, pour accomplir des missions non urgentes. ces soldats du feu sont devenus des soldats de la santé à force de pallier les lacunes de notre système de santé. Monsieur le ministre, à l'occasion du congrès de la fédération nationale à Vannes, il y a quelques jours, vous le rappeliez vous-même, il existe entre les Français et les sapeurs-pompiers une relation spéciale. Mais ces derniers n'en peuvent plus et notre modèle de sécurité civile est en danger. Les sapeurs-pompiers n'en peuvent plus de pallier toutes les sollicitations et de répondre à tous les défis : désertification médicale, réchauffement climatique, réorganisation et disparition des services publics dans les territoires ruraux. Toutes ces évolutions concourent à une situation malheureusement similaire à celles des urgences. Beaucoup de questions sont posées, mais peu de réponses leur sont apportées. Je n'évoquerai que quelques points. Concernant la directive européenne sur le temps de travail, aucune échéance n'a été donnée et aucune information n'est fournie. Nos volontaires demeurent dans l'expectative et s'inquiètent. La déclinaison des propositions de nature législative du rapport de la mission volontariat, ainsi que les nouvelles mesures de lutte contre les agressions- le Sénat fera prochainement des propositions à ce sujet -n'ont rationalisation du transport sanitaire héliporté. Enfin, en octobre 2017, le Président de la République appelait de ses voeux la mise en oeuvre d'un seul numéro d'appel d'urgence, le 112 : mise en oeuvre sans une régulation médicale devenue inopérante. Deux ans après, la France est encore à la traîne, alors que tous les autres pays européens ont depuis longtemps intégré cette nécessité. Monsieur le ministre, ma question est claire, et j'espère que votre réponse le sera tout autant votre gouvernement entend-il véritablement mettre en place une politique de sécurité civile ambitieuse et capable de faire face aux défis sociétaux et environnementaux à venir ?

et de l'alimentation. Hier après-midi, le débat en séance a porté sur la place déclinante de notre agriculture dans les marchés internationaux. Aujourd'hui, après une forte déprise- elle n'est pas récente -, notre agriculture n'occupe plus que 50 % de la superficie de notre territoire. Depuis plus de trois ans, une majorité de nos agriculteurs désespère. Leur revenu est de plus en plus bas, voire parfois inexistant. Des moyennes de revenus de 500 euros par mois sont la règle.

confrontés à une immense détresse, mettent fin à leur existence et plongent leur famille dans le deuil. Quel drame humain ! Que dirait-on d'une catastrophe qui, chaque année, ferait plus de 300 victimes ?

santé. Dans cette assemblée, au mois de juin dernier, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, nous débattions de l'obligation pour les étudiants de troisième cycle de médecine générale et d'autres spécialités d'effectuer leur dernière année en pratique ambulatoire, en autonomie, dans les zones caractérisées comme sous-dotées, et nous l'adoptions. La plupart d'entre nous savent combien les élus de territoires ruraux, mais aussi dans certaines villes, souffrent de la carence de médecins pour répondre aux problématiques de santé de leurs administrés. Je suis, par exemple, certain que, dans cette assemblée, nous avons, les uns et les autres, été interrogés par nos concitoyens sur leurs difficultés à trouver un médecin traitant. Cette mesure, madame la secrétaire d'État, est donc une bonne mesure, très concrète. Elle a été saluée par les associations d'élus, pour son caractère réaliste et pragmatique : non seulement elle instaure la présence d'internes en fin de formation dans des secteurs souffrant d'une offre de soins insuffisante, mais aussi elle facilite et incite l'installation de ces jeunes praticiens dans nos territoires.

l'engagement est pris de recruter 600 médecins salariés ou à exercice mixte ville et hôpital dans les déserts médicaux. Ma question est simple : comment comptez-vous procéder pour appliquer très rapidement ces mesures et de quelle façon envisagez-vous d'y associer les maires ?

nous accélérons le déploiement de 400 médecins généralistes, partagés entre la médecine de ville et l'hôpital, 200 dans les zones les plus modestes. S'agissant du développement des stages, la mesure a été adoptée, sur l'initiative de la dernière loi Santé. C'est une première réponse, efficace et pragmatique, à l'urgence territoriale. Nous nous inscrivons dans le calendrier que vous avez adopté. Nous souhaitons systématiser le stage ambulatoire en soins en autonomie supervisée pour les étudiants en dernière année d'internat à compter de 2021. dispositif seront définis par un décret, pouvant notamment ouvrir la possibilité d'une supervision à distance, afin de laisser davantage de souplesse dans l'organisation des terrains de stage.

sur la base des préconisations du rapport de la députée Anne Genetet. Nous avons ainsi remplacé la retenue à la source dérogatoire qui était appliquée à certains des revenus de source française, comme les traitements, salaires et pensions, par une retenue à la source de droit commun, déjà applicable aux mêmes revenus au-delà d'un certain seuil

Premièrement, l'application du droit commun, en lieu et place de la retenue libératoire, peut selon les cas se révéler plus ou moins avantageuse, en fonction, notamment, de la composition du foyer, de la part des revenus de source française ou de la nature des revenus. les contribuables non résidents ont toujours la possibilité, comme auparavant, d'opter pour l'imposition de leurs revenus au taux moyen, plutôt que la retenue à la source. Cette imposition consiste à appliquer, aux revenus de source française, le taux qui relèverait du barème de l'impôt sur le revenu- un barème progressif, donc -appliqué à l'ensemble des revenus mondiaux. ? La réforme, ajoutons-le, s'est accompagnée de nouveaux avantages pour les non-résidents, avec, notamment, la déduction des pensions alimentaires pour le calcul du taux moyen, ou encore l'allongement de cinq à dix ans

L'Unédic vient d'analyser les deux décrets réformant l'assurance chômage pris par le Gouvernement et le verdict est sans appel : les perdants seront nombreux ! Ce sont 1,3 million de personnes à la recherche d'un emploi qui vont voir leurs allocations de chômage baisser chômeurs sur dix ! Plus de 200 000 travailleuses et travailleurs sans emploi seront privés d'indemnités, soir 10 % des personnes concernées. En moyenne, l'Unédic estime que la baisse des allocations atteindra 19 %.

Les associations de personnes précaires et les centrales syndicales pressentent déjà que les premiers touchés seront les plus jeunes, qui enchaînent des contrats courts et de faibles salaires ; les plus fragiles.

Sa logique dissimule mal l'ambition d'économies budgétaires, au détriment de celles et ceux qui ont pourtant cotisé. Ma question est simple : qu'est-il prévu pour accompagner ces personnes, qui risquent de se retourner vers Pôle emploi ? Les agents craignent effectivement une montée d'agressivité et de colère,

Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d'honneur, d'une délégation de membres du Conseil national de Slovénie, conduite par M. Bojan Kekec, président de la commission des relations internationales et des affaires européennes. La délégation est reçue cette semaine au Sénat et en Seine-et-Marne par le groupe interparlementaire d'amitié France-Slovénie, présidé par notre collègue Colette Mélot. La visite en France de la délégation porte en particulier sur les thèmes de l'énergie et du climat et de l'économie circulaire. Elle sera aussi l'occasion d'évoquer les enjeux européens. Je forme le voeu que cette visite en France contribue à renforcer encore les liens qui unissent nos deux assemblées et nos deux pays. Mes chers collègues, en votre nom à tous et au nom du Sénat, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du Conseil national de Slovénie la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour

Michel Amiel, Julien Bargeton, Michel Dennemont, André Gattolin, Antoine Karam, Martin Lévrier, Frédéric Marchand, Thani Mohamed Soilihi, Georges Patient, Patricia Schillinger et Richard Yung figurent comme

lors du même scrutin, mon collègue Yves Daudigny et moi-même avons été notés comme ayant voté contre l'amendement n° 2 rectifié ; or nous avions l'intention de nous abstenir.

J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

C'est pour répondre à cette interrogation que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a lancé une mission relative à la sécurité des ponts. Je tiens à en remercier son président, Hervé Maurey, ainsi que mon collègue Michel Dagbert.

Après plusieurs mois de travaux, qui nous ont notamment permis de recueillir un grand nombre de témoignages d'élus locaux, les constats que nous avons présentés au début du mois de juillet dernier sont plutôt inquiétants.

En dix ans, le pourcentage des ponts gérés par l'État nécessitant un entretien sous peine de dégradation ou présentant des défauts a bondi de 65 % à 79 %. Plus de 700 ponts sont actuellement en mauvais état et exigent des travaux de réparation.

tout indique que ces infrastructures ont continué à se dégrader depuis, notamment du fait de la suppression, en 2014, de l'assistance technique que les services de l'État apportaient aux collectivités, de l'absence de politique généralisée de surveillance et d'entretien des ponts et de la dégradation de la situation financière des collectivités. D'après les experts que nous avons rencontrés, il est donc probable que, aujourd'hui, 18 % à 20 % des ponts des communes soient en mauvais état, soit plus de 16 000

ainsi à propos d'un ouvrage : « Pour le moment, la structure tient bien, mais il y aura des difficultés prochainement, vu la charge de matériel agricole. » Quant au maire du Poislay, dans le Loir-et-Cher, il explique que le pont reliant sa commune à celle de Droué exige des travaux très importants, car la réparation actuelle ne tiendra pas dans le temps ». Le mauvais état des ponts se traduit également par des restrictions de circulation et des fermetures, qui pénalisent les usagers dans leurs trajets quotidiens.

Plusieurs phénomènes expliquent que l'état des ponts se soit dégradé au cours des dernières années. Le premier, c'est vraisemblablement le vieillissement de ce patrimoine. Comme toutes Comme toutes les infrastructures, les ponts ont une durée de vie limitée. Or de nombreux ouvrages ont un âge avancé. Un quart des ponts gérés par l'État été construits entre 1950 et 1975. Ils sont ou seront donc prochainement en fin de vie. De même, l'âge du patrimoine des ponts des communes dépasse souvent cinquante

car elles ne disposent ni de l'expertise en interne ni des ressources financières suffisantes pour solliciter une expertise privée. Le diagnostic de l'état d'un pont et les travaux d'entretien et de réparation peuvent représenter un coût important pour elles.

fermés à la circulation depuis 2014 en raison de leur mauvais état. Les travaux de réhabilitation sont estimés à 1 million d'euros pour chacun d'eux, alors même que le budget annuel de ces communes n'excède pas les 3 millions d'euros ... Ce constat nous a conduits à faire plusieurs propositions. La première de ces propositions est d'ordre financier. Il ne faut pas se leurrer : sans moyens supplémentaires, il est évident que nous ne pourrons pas enrayer la dégradation de l'état de nos ouvrages d'art.

la gestion patrimoniale des ponts, en particulier en améliorant la prise en compte des dépenses d'entretien de ces ouvrages dans la comptabilité publique, en renforçant la connaissance de ce patrimoine par un système d'information géographique national

-certaines d'entre elles méconnaissent l'état de leurs ponts, voire leur nombre, ne sont pas équipées pour en assurer la gestion et se heurtent à des difficultés financières. Pour répondre à ces problématiques, la mission, dont je salue le travail, a formulé un certain nombre de recommandations.

à l'initiative de cette mission consacrée à la sécurité des ponts, ainsi que les rapporteurs, MM. Patrick Chaize et Michel Dagbert. Je mesure l'urgence de la situation et souhaite que nos propositions soient rapidement suivies d'actions. Le constat est alarmant : nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe comme l'effondrement du pont Morandi. La situation est d'autant plus grave qu'elle est complexe. En effet, d'une part, la gestion du réseau se partage entre l'État et les collectivités locales d'autre part, les collectivités ne sont financièrement pas en mesure de prendre en charge la rénovation et l'entretien des 90 % du réseau qui leur échoient.

Quand ils surviennent, c'est bien souvent qu'il est déjà trop tard. Il s'agit de désordres visibles, évidents, signalés par les riverains ou les usagers, et les travaux afférents sont forcément coûteux. Participant à cette mission d'information et revenant sur ma propre expérience, je me suis demandé pourquoi, sur ce sujet particulier, nous pratiquions presque tous la politique de l'autruche. En effet, pourquoi pensons-nous à surveiller nos toitures, nos chaudières, nos gouttières, et oublions-nous nos ponts ? Pourquoi faisons-nous comme si les ponts étaient éternels ?

et 5 000 euros par ouvrage -, recourir forcément à une entreprise spécialisée qui saura respecter des procédures désormais complexes. Je tenais donc, monsieur le secrétaire d'État, à attirer votre attention sur ce point : l'entretien courant n'est plus possible au-dessus d'un cours d'eau.

Bien des collectivités manquent d'une connaissance exacte des transferts de compétences qui se sont opérés au cours du temps. Les ouvrages se dégradent ; s'ils sont anciens, aucune convention n'établit clairement le partage des charges et responsabilités- Mme Assassi a parlé longtemps de la loi Didier. Vous avez dit que le recensement qui était prévu pour le 1 janvier

le rapport remis par notre mission a mis en exergue un état de vétusté inquiétant de nos ouvrages d'art, dont l'état structurel, pour 25 000 d'entre eux, pourrait mettre en péril la sécurité des usagers. Les collectivités territoriales sont particulièrement affectées, puisque ce problème touche 20 % des ponts relevant des communes ou des intercommunalités. Parmi ces dernières, les plus petites sont largement démunies : pas d'ingénierie technique, pas de ressources budgétaires ni d'assise financière suffisante pour obtenir les prêts permettant de conduire les travaux. J'en veux pour preuve la situation d'une commune de mon département qui, avec ses 2 500 habitants, et après avoir déjà financé une expertise à hauteur de 6 000 euros, devrait supporter une dépense de l'ordre de 700 000 euros pour la remise en état d'un ouvrage d'art rétrocédé par VNF sans que la ville n'ait rien demandé. Le plan Marshall pour les ponts sollicité par la mission devient, dans ce contexte, une absolue nécessité- je pense en particulier à la création d'un fonds d'aide aux collectivités territoriales doté de 130 millions d'euros par an sur une période de dix ans.

ne saurions laisser dire qu'un simple jeu de vases communicants suffirait à répondre à de tels enjeux. Nous demandons non pas une réorientation de crédits, mais bien la mobilisation d'une enveloppe nouvelle, et espérons que le débat prochain sur le projet de loi de finances sera l'occasion pour l'État de prouver qu'il a pris la pleine mesure de la situation. La parole

d'État, mes chers collègues, chacun garde en mémoire les images terribles de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc qui, le 24 mars 1999, avait suscité une très grande émotion en France, ou celles de l'effondrement du pont Morandi de Gênes, l'année dernière. Hier encore, un pont long de 140 mètres s'est écroulé à Taïwan. Ces infrastructures sont donc un enjeu majeur de sécurité pour les usagers.

dédié au renforcement de la sécurité des 700 ouvrages que compte son territoire et qui sont régulièrement suivis. Mais ce sujet pose des difficultés pratiques lorsque les ponts enjambent des voies SNCF ou des voies d'eau. Ces difficultés sont de deux ordres : premièrement, la responsabilité relative à l'entretien voire à la reconstruction de l'ouvrage

Je prendrai rapidement l'exemple du pont Saint-Ladre, à Crépy-en-Valois. Construit en 1929 par la compagnie des chemins de fer, il appartient au gestionnaire de la chaussée, mais son entretien doit être assuré par la SNCF. En 2008, la SNCF inspecte le pont. En 2013, le département intervient auprès de la SNCF pour connaître connaître l'état de la structure, et celle-ci fait savoir qu'elle envisage la reconstruction du pont, pour finalement abandonner cette idée en 2015. En 2016, le département introduit un référé pour que la justice statue sur la responsabilité. Un expert est désigné, qui conclut à l'interdiction du passage des poids lourds. Depuis, c'est le statu quo.

les objets technologiques comme des systèmes complexes, dont les éléments, en interaction dynamique les uns avec les autres, pouvaient entrer en résonance jusqu'au dépassement des limites de rupture. D'où l'importance de l'analyse, de l'expertise, de la vigilance et de la surveillance, qui permettent, le cas échéant, de déclencher les interventions prédictives ou curatives les plus appropriées. de nos collectivités territoriales, qui gèrent désormais à elles seules plus de 90 % du réseau routier français, le rapport met en évidence divers constats. Le transfert des compétences qui s'est opéré s'agissant notamment de la voirie et des ouvrages d'art ne s'est pas toujours accompagné des plans de récolement des ouvrages et de toute la documentation technique associée. Ceux-ci ont souvent été égarés ou se sont avérés incomplets, à moins que l'évolution des interventions sur les ouvrages

un futur désirable, dans la mesure où des expérimentations existent déjà. En général, celles-ci portent sur des objets qui ont présenté des fragilités, des difficultés ou des dysfonctionnements particuliers,

: celui du pont de Petite-Rosselle. Cet ouvrage construit au milieu du XIX siècle pour les besoins de l'exploitation charbonnière et permettant la liaison routière entre les communes de Petite-Rosselle et de Forbach est aujourd'hui dans un état de délabrement tel qu'il est urgent de procéder à sa reconstruction. L'État en étant propriétaire- toutes les recherches effectuées par la commune l'attestent -, il est normal qu'il assure la charge de cette reconstruction. Mme la ministre Élisabeth Borne en était d'ailleurs entièrement d'accord puisque, le 19 mars 19 mars dernier, en séance publique, elle déclarait : « le pont de Rosselmont appartient sans ambiguïté à l'État, eu égard à la reprise par celui-ci du patrimoine des houillères. [ ...] Je confirme qu'il appartient à l'État, dans le cadre de sa mission de gestionnaire de l'ancien patrimoine des houillères, de remettre ce pont en état. Les travaux à cette fin vont être programmés. » Par conséquent, vous comprendrez la perplexité du maire de Petite-Rosselle

lire l'allemand et même la Elle n'a trouvé aucune trace, ni directe ni indirecte, qui pourrait laisser penser qu'elle a pris part, de près ou de loin, à la construction de ce pont.

Lefèvre. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, dans le cadre de la loi Didier du 7 juillet 2014, l'État a procédé à un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies publiques interrompues par une nouvelle infrastructure de transport pour lesquelles aucune convention de répartition des charges n'existait avant l'entrée en vigueur de cette loi. Parmi ces ouvrages, l'État identifiera ceux dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifieront la conclusion d'une convention dans les conditions définies par la loi. Or bon nombre d'ouvrages SNCF affectant des routes départementales ou voies communales de mon département, l'Aisne, ne figurent pas dans la liste provisoire qui a été publiée par l'État au mois d'août Lors de leur reconstruction, ces ouvrages ont en effet donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de récolement fixant la répartition des charges d'entretien des ouvrages auxquels le Conseil d'État a admis une valeur conventionnelle. Cependant, ces procès-verbaux ne contiennent aucune disposition en matière de répartition des charges de grosses réparations, de démolition et de reconstruction des ouvrages, si bien que le gestionnaire de la voie portée ne dispose d'aucun moyen de recours à l'égard de l'exploitant de la nouvelle infrastructure en dehors des opérations d'entretien courant. Si seuls les ouvrages figurant sur la liste qui sera définitivement arrêtée par l'État pourront faire l'objet d'une convention nouvelle, le problème est donc le suivant : la question des interventions majeures sur les ouvrages non recensés restera entière pour les collectivités gestionnaires

notamment par les établissements publics que sont le Cérema et l'Ifsttar, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Le rapport d'information a mis en avant les carences de la politique de gestion des ponts menée par l'État, s'agissant tant des méthodes d'évaluation des ponts que de leur entretien. Nous connaissons pourtant l'importance de la mise en oeuvre d'une politique de surveillance et d'entretien pour la sécurité des ouvrages d'art. Alors que l'expertise des établissements publics précités paraît de plus en plus indispensable pour effectuer une analyse des risques et réaliser les travaux d'entretien nécessaires, les moyens qui leur sont accordés sont en constante diminution. Les effectifs du Cérema n'ont en effet cessé de baisser, la réduction annuelle du plafond d'emploi étant de l'ordre de 4 % ces dernières années. Cette baisse des effectifs, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas sans conséquence sur son activité ; le Cérema indique d'ailleurs que la mise en oeuvre de sa stratégie d'évolution relative à la gestion du patrimoine est entravée notent les auteurs du rapport, cette situation pourrait non seulement réduire ses capacités d'intervention, mais aussi entraîner une perte de compétences de l'établissement.

de répondre aux interrogations légitimes de nos concitoyens. Son excellent travail sur la sécurité des ponts a mis en exergue les nombreuses lacunes de la France, en particulier l'absence de contrôle effectif, faute d'un recensement exhaustif de nos ouvrages. Selon la mission- cela a été dit -, 25 000 ponts sont en mauvais état structurel et posent, à ce titre, des problèmes de sécurité pour les usagers. Il y a donc urgence à agir. Le projet de loi d'orientation des mobilités était justement l'occasion de répondre à cette urgence en permettant à l'État de soutenir financièrement les collectivités au travers des financements alloués à l'Afitf. Nous avions anticipé, au Sénat, en inscrivant dans le texte qu'« en partenariat avec les collectivités territoriales, premiers gestionnaires de ce patrimoine, et dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, l'État accompagnera l'inventaire, la surveillance, l'entretien et, le cas échéant, la réparation de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour l'attractivité française et présentent aujourd'hui des risques de sécurité mal connus. de sécurité mal connus. » Je regrette que cette solution n'ait pas été retenue par l'Assemblée nationale, qui lui a préféré un simple accompagnement logistique sans aucune garantie financière. suite de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc en 1999, l'État a pourtant débloqué, via l'Afitf, des fonds exceptionnels de 1,2 milliard d'euros sur onze ans entre 2007 et 2018, afin de financer la mise en sécurité des tunnels de notre réseau routier. La mission d'information démontre bien que nous ne sommes pas à l'abri d'un accident qui toucherait nos ponts les plus vétustes. Faut-il prendre le risque d'attendre un drame en France pour que nos ponts bénéficient des fonds nécessaires à leur mise en sécurité ? Entendez-vous, monsieur le secrétaire d'État, reprendre les propositions formulées par le Sénat dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités ou valider la création du fonds préconisé par la mission ?

mauvais état » ne veut pas dire « dangereux ». On estime que 6 % des ponts en France sont en mauvais état, c'est-à-dire qu'ils présentent des dégradations nécessitant un entretien à un horizon plus ou moins lointain, mais en général relativement proche. Les ponts qui sont jugés dangereux sont interdits à la circulation.

cette fameuse trajectoire qui est portée à 120 millions d'euros par an à compter de 2023 ; d'autre part, les financements nouveaux qui seront le fruit des discussions actuelles sur les ouvrages dits de « rétablissement » et dont

de la part de VNF. Mme la ministre m'avait confirmé par écrit que ce pont faisait bien partie de l'inventaire des ouvrages concernés par la loi Didier. Au mois de juin dernier, nous avons organisé une rencontre

que l'ouvrage en question figurera dans le recensement des ouvrages d'art dits « de rétablissement » en vertu de la loi Didier. Une réunion s'est bien tenue le 7 juin 2019, qui pose les grandes bases de ce que sera éventuellement la convention de répartition des charges.

Les autoroutiers sont dans une situation un peu différente de ce point de vue. Je m'interroge néanmoins sur le risque d'un accident et d'une crise qui viendraient clarifier la situation et accélérer les choses. C'est une situation que nous ne souhaitons absolument pas. Vous pourrez compter sur

la mission d'information sur la sécurité des ponts souligne la nécessité d'une gestion patrimoniale des ponts. Nous avons tous des exemples, dans nos territoires respectifs, de ponts vieillissants, insuffisamment entretenus, fermés à cause d'un péril imminent. Souvent, il s'agit d'ouvrages majeurs, alors même que nous n'avons aucune idée précise de l'état des petits ponts fortement endommagés. Un exemple emblématique dans le département de la Loire-Atlantique est le pont de Saint-Nazaire, point stratégique majeur reliant la Bretagne à la

Près de 30 000 véhicules le franchissent chaque jour. Le département de Loire-Atlantique, chargé de son entretien, doit faire face aux besoins permanents de travaux de consolidation. Le béton est dégradé par les embruns maritimes. Les campagnes d'entretien sont d'entretien sont longues et coûteuses pour les collectivités territoriales : de 2010 à 2014, le pont a fait l'objet de 20 millions d'euros de réparation sur sa partie sud et de 8 millions d'euros sur sa partie nord en 2018. Il a même fallu prévenir l'affaissement des travées en renforçant des poutres en béton. Tous les trois ans, des spécialistes auscultent sur plusieurs mois les semelles et les fondations immergées des piles. Je viens d'évoquer la situation du plus long pont de France, lui-même touché par les outrages du temps. Mais, à côté des ouvrages de premier ordre, combien de petits ponts subissent des désordres dans l'indifférence ? On estime à plus de 200 000 ces ouvrages qui structurent les voies de nos communications quotidiennes. La mission d'information souhaite intégrer dans les budgets des collectivités locales les dépenses de maintenance des ouvrages. Nous attendons un signal fort de l'État, car un tiers des ponts sous sa responsabilité sont en mauvais état.

Ma question sortira du sujet des ponts, mais porte néanmoins sur la sécurité des structures. À la suite d'un accident tragique survenu dans mon département- la chute d'un balcon à Angers en 2016 -, j'avais attiré l'attention du Gouvernement sur la nécessaire certification des armatures du béton. Le béton armé est le matériau de construction le plus utilisé en France. L'incorporation d'armatures est indispensable au renforcement de la solidité de l'ouvrage, mais des armatures de mauvaise qualité ou une pose incorrecte peuvent avoir des conséquences dramatiques.

concernent les balcons. Néanmoins, dans 15 % des dossiers, un défaut sur la structure des balcons a été relevé, avec un placement défaillant ou une mauvaise mise en oeuvre du béton. L'étude propose des perspectives d'amélioration, avec l'instauration d'audits ou des contrôles de la disposition des armatures. Mais qu'en est-il de la certification des armatures ? Plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, ont introduit une certification obligatoire pour les entreprises fabricant ou mettant en oeuvre ces armatures. L'Association française de certification des armatures du béton alerte les pouvoirs publics depuis plusieurs années sur la nécessité de recourir à des armatures de qualité et à des entreprises de

fassiez une réponse différée. La parole est à M. le secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous me surprenez en flagrant délit d'incompétence sur le sujet. Je vais me rapprocher de mon collègue ministre de la cohésion des territoires pour avoir accès au dossier et vous adresser une réponse écrite, qui sera certainement plus précise et plus intéressante que celle que je pourrais vous faire ici

Comme souvent, il aura fallu attendre une terrible catastrophe pour mettre en évidence le vieillissement de ce type d'infrastructures et se pencher, par voie de conséquence, sur leur état en France. Dès lors, cela nous renvoie évidemment au défi lié à leur entretien. Je tiens à cet instant à remercier nos collègues sénateurs Patrick Chaize et Michel Dagbert pour avoir conduit ce travail particulièrement utile avec la mission d'information sur la sécurité des ponts. Bien entendu, plusieurs ingénieurs tirent la sonnette d'alarme et appellent à investir davantage. Mais la véritable question, comme d'habitude, est : « Qui va payer ? Premier constat, en France, ce sont les collectivités territoriales qui sont en première ligne. Il s'agit d'une spécificité française ! Les communes et les départements gèrent près de 90 % de ces ouvrages d'art. Je suis marqué par le désarroi des élus locaux qui gèrent des communes de taille modeste. Aujourd'hui, 20 % des ponts communaux présenteraient une structure altérée ou gravement altérée, soit un total de 16 000 ponts potentiellement dangereux. Or les communes manquent de ressources financières pour régler ce problème.

bâtiments communaux, une église du XVI siècle, 56 kilomètres de voirie, 100 kilomètres de canalisations, trois ponts et un viaduc avec une dotation globale de fonctionnement en retrait de 650 000 euros sur quatre Ma question est simple, monsieur le secrétaire d'État : la création d'un fonds d'aide spécifique aux collectivités locales est-elle envisageable afin de leur permettre d'effectuer un suivi patrimonial des ponts et d'entreprendre les travaux nécessaires à leur sécurisation ? La parole est à M. le

La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-338 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 29 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Jean-Pierre Farandou aux fonctions de président du directoire de la SNCF.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, parce qu'elle concentre de forts enjeux stratégiques, éthiques et économiques, l'émergence de l'intelligence artificielle est communément qualifiée de quatrième révolution industrielle. Aussi, le RDSE a souhaité que le Sénat en débatte ce soir. J'en profite pour saluer les travaux du groupe de suivi de notre assemblée qui s'est emparé de ce sujet dès 2017. Si l'intelligence artificielle fut pour la première fois évoquée en 1956 dans le cadre d'une conférence universitaire aux États-Unis, ce sont les recherches technologiques les plus récentes qui permettent son développement fulgurant. Je ne m'attarderai pas sur sa définition qui, vous le savez, interroge souvent, tant cet outil est « disruptif ». Pour faire simple, je dirais qu'il s'agit de seconder l'intelligence humaine pour augmenter celle-ci ... La compilation de données du big data combinée à la puissance de calcul ouvre des horizons incroyables pour effectuer des fonctions, pas forcément toujours mieux que le ferait un homme, mais en tout cas beaucoup plus rapidement. Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle a investi de nombreuses applications qui commencent à envahir notre quotidien : voitures autonomes, diagnostics médicaux, finance algorithmique, robots industriels, jeux vidéo ... Ces applications ne sont que le début d'un développement irréversible, une tendance qui charrie également nombre de craintes et de phantasmes. Je balaierai tout de suite celui de la perte du contrôle de l'intelligence artificielle, qui conduirait la machine à échapper à son créateur, une situation largement véhiculée par des oeuvres de fiction littéraire ou cinématographique. Même si je n'ignore pas la lettre ouverte cosignée en 2015 par 700 chercheurs de renom alertant l'opinion sur l'hypothèse d'une « intelligence artificielle malveillante ou trop autonome je pense qu'il est préférable de croire à la possibilité d'en fixer les limites, d'en encadrer les usages. Raisonner autrement nous obligerait à renoncer à une partie du potentiel offert par l'intelligence artificielle et à laisser des États moins scrupuleux s'en emparer complètement. Par ailleurs, relativisons la vision d'une intelligence artificielle triomphante. En effet, si la machine peut atteindre une puissance extraordinaire pour la réalisation de nombreuses tâches, il lui manquera toujours ce qui fait notre singularité et notre supériorité sur elle en tant qu'êtres vivants : l'intuition et l'imagination. Cette inquiétude pose en tout cas le débat des enjeux éthiques. Je m'arrêterai un instant sur la question de la protection des données, la matière première qui alimente l'intelligence artificielle. Notre pays est particulièrement soucieux de la protection des données, tout comme l'Union européenne, qui dispose d'un marché de 500 millions de consommateurs qu'elle doit impérativement protéger. C'est tout le sens des dernières législations adoptées par l'Union, au premier rang desquelles le règlement relatif à la libre circulation des données à caractère non personnel, la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public, ou encore les règles relatives à la cybersécurité. L'Europe s'est dotée d'un véritable cadre juridique, que l'on ne peut qu'applaudir. Au-delà de la protection des données, il doit aussi être question de responsabilité, de transparence des algorithmes et d'information sur les décisions sous-jacentes aux applications. L'intelligence artificielle doit également être inclusive, et ce à double titre : n'oublier personne pour les bénéfices qu'elle apporte, et protéger tout le monde des bouleversements qu'elle pourrait induire sur le plan sociétal. en particulier à l'organisation du travail, qui pourrait être impactée à la fois négativement et positivement. Dans ces conditions, mes chers collègues, et comme le souligne très clairement le rapport intitulé, remis au Gouvernement par Cédric Villani et rendu remis au Gouvernement par Cédric Villani et rendu public l'année dernière, doit-on autoriser l'accès aux données européennes à des entreprises qui ne seraient pas implantées en Europe et qui ne se plieraient donc pas à nos principes éthiques ? Cette réserve ? Cette réserve s'impose en raison de la domination des Gafam sur la récupération de données et, plus globalement, en raison de la compétition entre la Chine et les États-Unis qui prend en étau l'Union européenne. Nous savons, s'agissant des États-Unis, que les Gafam leur donnent un avantage considérable. Leur avance en termes de collecte des données, de matériel de pointe et de recherche sera- soyons lucides -difficilement rattrapable. Les investissements Les investissements qu'ils consacrent à l'intelligence artificielle, cumulés à ceux que les pouvoirs publics américains injectent de leur côté par le biais de leurs grandes agences, leur confèrent un leadership indétrônable pour les années qui viennent. Quant à la Chine, elle ambitionne de contester ce leadership en investissant chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, quel est le niveau de l'ambition européenne ? En avril 2018, la Commission a jeté les bases d'une stratégie sur l'intelligence artificielle ayant pour but d'augmenter les investissements publics et privés, afin qu'ils atteignent au moins 20 milliards d'euros par an au cours des dix prochaines années.

avec le rachat de l'entreprise anglaise DeepMind par Google et de l'allemande Kuka par un groupe chinois. En février dernier, le Conseil européen a confirmé les propositions de la Commission visant à faire de l'Europe un acteur de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle, et souhaité que les États membres investissent dans tous les secteurs économiques. Soit ! Mais, à cet égard, compte tenu des besoins colossaux de financements, il me semblerait pertinent que chacun des États membres s'emploie plutôt à performer sur un segment, tandis que l'Union européenne positionnerait de son côté des champions européens sur divers secteurs par le biais des « projets importants d'intérêt européen Piiec. Parmi les secteurs que notre pays doit privilégier, je pense à celui de la santé, dont la croissance du volume de données créées sera la plus forte d'ici à 2025. Dans ce domaine, compte tenu de son système de protection sociale, la France dispose d'un atout de taille : une centralisation forte des données par l'administration. Nous avons par ailleurs intégré le le RGPD, dans notre législation, ce qui doit permettre de garantir la sécurité de l'exploitation de données médicales, des données qui sont bien entendu Je citerai également le secteur de la sécurité, comme l'a préconisé la ministre des armées à Saclay le 5 avril dernier. Il s'agit là, pour des raisons stratégiques évidentes, de nous appuyer sur l'intelligence artificielle pour conserver notre supériorité opérationnelle. Dans le monde numérique Dans le monde numérique qui nous attend, le principal défi est de pouvoir conserver notre souveraineté, qu'elle soit économique, politique ou stratégique. Le maintien de notre indépendance par le développement de nos propres outils d'intelligence artificielle est le gage de la protection des libertés de nos concitoyens, de notre territoire et d'une transformation douce de notre économie pour réaliser une répartition juste de la valeur au bénéfice de tous. Ce défi, vous l'aurez compris, impose la mobilisation de moyens considérables afin de nous permettre d'agir en amont plutôt que de subir. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous remercie d'avoir été attentifs à mon intervention, qui n'a pas été rédigée à la plume Sergent-Major, mais qui n'est pas non plus le fruit d'un algorithme, bien heureusement. La parole est à M. le secrétaire

clés font aujourd'hui l'objet d'une bataille technologique mondiale, dominée par les Américains et les Chinois. La question qui se pose à nous est donc celle de la capacité de l'Europe à faire émerger qui soient à la hauteur de Google ou de Facebook, dont je rappelle qu'ils ne sont pas des spécialistes de l'intelligence artificielle : au début, Google était un moteur de recherche et Facebook un réseau social. Mais l'économie mondiale est ainsi faite que ces groupes grossissent, se développent et dégagent des marges considérables

Dans certains domaines, en effet, nous allons voir arriver des applications ou des sociétés dont les produits seront meilleurs que ceux de nos entreprises, parce qu'ils auront été développés grâce à des bases de données incontrôlées.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Face à l'attractivité et à la prédation de ces conglomérats supranationaux, quelle est la stratégie du Gouvernement pour enrayer la fuite des cerveaux de la recherche française ? fondamentale. Si vous ne parveniez pas à développer une telle stratégie, nous perdrions à très court terme toutes les capacités intellectuelles de notre pays au profit des Gafam. Vous avez

de concentrer une partie de nos forces sur quatre hubs de recherche- Paris, Grenoble, Toulouse et Nice -et de créer, dans ces cadres-là, un écosystème

recherche. Très bien ! La parole est à M. Joël Guerriau. Je tiens à saluer l'initiative de nos collègues du RDSE d'ouvrir le débat sur les enjeux économiques et stratégiques de l'intelligence artificielle. Le groupe Les Indépendants avait eu l'occasion, à l'automne 2017, d'interpeller le Gouvernement sur cette problématique majeure du XXI siècle, dans le cadre d'un débat parlementaire orienté sur le rôle que la France et l'Europe peuvent encore espérer jouer dans cette course à l'innovation. Le constat que nous faisions n'était guère réjouissant. Deux ans plus tard, ces craintes n'ont pas disparu ; au contraire, elles se sont même renforcées. Et pour cause : preuves ne cessent de s'accumuler qui démontrent qu'il s'agit bel et bien d'une nouvelle révolution technologique. Elle percutera de plein fouet notre modèle social ainsi que nos modes d'organisation. L'intelligence artificielle recourt à des algorithmes pour reproduire des processus cognitifs humains. D'où le sentiment de dépossession que nous éprouvons souvent face à ses utilisations toujours plus diverses. Les robots imitent de mieux en mieux les humains, au point qu'il est devenu monnaie courante de les confondre, tantôt en écoutant la réponse pleine d'humour d'un assistant vocal, tantôt en lisant un message personnalisé prérédigé par un téléphone dit « intelligent Le risque existe de voir émerger à grande échelle de nouveaux réseaux de crime organisé qui utiliseraient l'intelligence artificielle pour mieux tromper particuliers et entreprises. La menace existe déjà. C'est notamment le cas avec les image les image et voix humaines sont copiées et l'identité est détournée pour diffuser de fausses informations. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous confirmer que les services de l'État agissent pour faire face à cette nouvelle forme de délinquance et de piratage ? Quelles mesures sont prévues pour cibler et punir ces délinquants et ces criminels

La Chine a créé un « cybermur » pour imposer un contrôle social de sa population, en combinant réseaux sociaux, caméras à reconnaissance faciale et intelligence artificielle. Elle utilise l'intelligence artificielle à des fins de contrôle social à très grande échelle,via un système algorithmique de reconnaissance faciale. Chaque citoyen et chaque entreprise disposent d'un capital initial de mille points. En fonction de leurs comportements et fréquentations, ils gagnent ou perdent des points. « Les mauvais citoyens » sont sujets à des restrictions médicales, d'accès à l'emploi ou à des interdictions de déplacement. Cela peut également se traduire par des traitements d'humiliation sociale, par l'affichage sur la voie publique et sur écran géant du portrait d'un passant en retard de paiement ou ayant jeté un mégot dans la rue. Cette dictature 5G utilise ses Routes de la soie pour tenter de prendre subrepticement le contrôle de pays en liant son aide à la signature de contrats de fourniture d'équipements technologiques. Un tiers des pays du monde ont d'ores et déjà signé des partenariats avec les entreprises chinoises pour leur acheter ces technologies.

exemple ? Notre pays dispose-t-il d'un plan pour nous protéger des pratiques intrusives chinoises, susceptibles de menacer à terme nos libertés ?

puisque nos entreprises ne peuvent pas garantir à certains citoyens chinois la protection de leurs données et une approche démocratique, il faut appliquer le principe de réciprocité à l'envers : ce qui est interdit pour nos entreprises doit être interdit pour les entreprises chinoises au sein de l'Union européenne. Je pose la question : dans quel monde voulons-nous vivre demain ?

C'est précisément l'un des axes de la stratégie européenne pour l'intelligence artificielle que propose la Commission européenne, avec l'ambition qu'y soient consacrés pas loin de 20 milliards d'euros chaque année à partir de 2021. La France doit saisir cette initiative européenne et se positionner en leader de l'intelligence artificielle en Europe avec l'Allemagne. Car, face aux géants américains et chinois, ce n'est qu'à l'échelle européenne que pourra se déployer une stratégie globale prenant en compte les dimensions non seulement scientifique et économique, mais aussi éthique et sociétale de cette nouvelle forme d'économie, et capable de faire prévaloir une approche fondée sur la transparence et la confiance. Dans un rapport publié en janvier 2019, la commission des affaires européennes appelait à utiliser tous les moyens pour combler notre retard. Sur ce fondement, le Sénat a recommandé dans une résolution européenne de mars dernier que l'intelligence artificielle puisse faire l'objet d'un projet important d'intérêt européen commun, comme ce fut le cas avec succès pour la micro-électronique. Ce mécanisme, prévu par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permet, sous certaines conditions, le versement d'aides financières de la part de plusieurs États membres. Ainsi, nous pourrons construire cet « Airbus de l'intelligence artificielle » que les ministres français et allemand de l'économie appelaient encore de leurs voeux il y a quelques jours. Il en résulterait des effets d'entraînement positifs pour l'ensemble des vingt-sept États membres. Monsieur le secrétaire d'État, comptez-vous porter comptez-vous porter cette ambition devant le Conseil pour contribuer, au-delà des coopérations bilatérales que nous saluons, à la mise en place d'une véritable stratégie industrielle européenne en faveur de l'intelligence artificielle ? Très bien M. le secrétaire d'État. Le projet que vous évoquez est au coeur de la volonté commune de Bruno Le Maire et de Peter Altmaier de travailler à la souveraineté européenne en faisant émerger un certain nombre de champions dans des domaines particulièrement stratégiques pour la souveraineté européenne comme l'intelligence artificielle. Vous avez cité, monsieur le sénateur, l'« Airbus de l'intelligence artificielle », évoqué par les deux ministres, mais on peut également penser au projet

réalité sémantiquement plus large. Ma question portera sur les conséquences de cette technique sur le travail et l'emploi. Nous le constatons aujourd'hui avec les travailleurs du clic et de la nouvelle industrie des plateformes, le monde du travail est peu préparé à l'économie du numérique qui émerge sous nos yeux partout dans le monde. Il est très difficile d'évaluer les conséquences du développement de l'intelligence artificielle, de l'automation et de la robotique, notamment en termes de solde des emplois qui en résultera.

appelle à une réflexion sur les modes de complémentarité entre l'humain et l'intelligence artificielle, une complémentarité non aliénante, mais source de progrès pour l'humanité et prenant en compte la dimension écologique de l'économie nouvelle émergente. Dans ce contexte, quelles initiatives et démarches structurées le Gouvernement compte-t-il prendre pour refondre le pacte social et républicain, d'ores et déjà affecté par ces nouvelles formes de travail ? Dans un ouvrage récent, la sociologue Dominique Méda relève que « le capitalisme de plateforme participe de l'émergence de formes renouvelées, voire exacerbées, de sujétion du travailleur ». La proposition intéressante de Cédric Villani de créer un « lab public de la transformation du travail » retient-elle votre intérêt pour articuler ces grandes transformations sociétales avec les politiques publiques, qui doivent les prendre en compte et même les anticiper ? La parole est

qu'il faut définir un cadre national, mais que les choses se feront par bassin d'emploi. C'est autour de Perpignan, de Lille, que les employeurs, les organisations syndicales, les collectivités territoriales, Pôle emploi et l'État doivent travailler pour identifier combien de

pays dans le monde. La parole est à M. Jean-Yves Roux. Les usages de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui y président sont multiples, croissants et, dans bien des cas, invisibles et incompréhensibles pour le commun des mortels. Parmi les usages les plus emblématiques, je citerai les fils d'actualité des réseaux sociaux. Or ces réseaux constituent pour les jeunes de 15 ans à 34 ans les vecteurs d'information principaux dans plus de 70 % des cas. Les algorithmes qui régissent les réseaux sociaux et les mécanismes de traitement des données associées nourrissent tous les fantasmes et autorisent des manipulations d'opinion. reprendre un propos de Tristan Mendès France, maître de conférences à la Sorbonne, spécialiste des nouveaux médias, « les algorithmes accentuent, non pas ce qui est vrai, mais ce qui est choquant, ce qui est clivant Le rapport de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de décembre 2017 sur les algorithmes à l'heure de l'intelligence artificielle posait déjà la question en ces termes : comment permettre à l'homme de garder la main ?

le débat démocratique, la Constitution, la République posent des règles- l'égalité hommes-femmes, des principes non discriminatoires, le respect de la vérité -, la fabrique de l'opinion pour les jeunes générations s'opère très majoritairement dans un espace dérégulé, international, dans lequel la réalité peut être distendue.

pour chaque personne et pour chaque profil. Ensuite se pose la question de la régulation, qu'il ne faut d'ailleurs pas prendre uniquement dans le sens de l'information. La proposition de loi de la députée Laetitia Avia arrive au Sénat, et nous aurons l'occasion de débattre des contenus haineux.

l'un de l'autre. En réalité, un grand nombre de dispositifs utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour accompagner au quotidien nos concitoyens. L'intelligence artificielle se positionne ainsi comme un vecteur innovant pour rendre l'administration française plus proche des besoins des usagers, plus efficace, plus efficiente et tournée vers l'avenir. Porteuse d'opportunités nouvelles, elle favorise le recentrage des agents publics sur leur coeur de métier, sans diminuer le contact humain. Monsieur le secrétaire d'État, je connais votre implication sur le sujet. Aussi, pouvez-vous nous dire quelles sont les prochaines étapes prévues par le Gouvernement pour accompagner la transformation de notre administration ?

présentait les grandes lignes de sa stratégie de recherche en matière d'intelligence artificielle, à laquelle seront consacrés 665 millions d'euros d'ici à 2022. Le Gouvernement entendait notamment augmenter les financements de doctorants en intelligence artificielle et le nombre de ces derniers, qui était d'environ 250. Il projetait également de créer 40 chaires via un appel à candidatures national et international. Sur ce point précis, où en sommes-nous ?

nous sommes pleinement conscients que des machines autonomes pourraient demain prendre le contrôle de nos existences, utiliser nos données comme bon leur semble pour, par exemple, nous exclure de la société ou renforcer une élite. Les machines ont désormais des capacités « d'apprentissage profond elles peuvent tirer des points communs ou des règles statistiques d'une immense quantité de données. Elles reconnaissent ainsi une image ou un son, orientent un véhicule ou une personne. Dans ces conditions, pourquoi ne pas s'engager davantage ? Les Français le comprendraient aisément et rejoindraient M. Villani, notre médaille Fields, quand il dit : « Il [ ...] un travail d'éducation à faire pour défendre la responsabilité humaine, éviter que des algorithmes surestimés ne renforcent des discriminations, et définir le meilleur partage des tâches entre humains et machines.

Le programme national de recherche présenté par le Président de la République a quatre objectifs : constituer un réseau national attractif pour les acteurs de la recherche en intelligence artificielle ; mettre en place des outils pour réaliser cette recherche académique ; recourir à des mesures incitatives pour développer la recherche partenariale entre le privé et le public ; et, enfin, augmenter le nombre de doctorants et de chaires- vous avez cité les sommes que nous y investissons. La mise en oeuvre du plan avance très bien. Les instituts

Elle a pour particularité, en matière de défense, d'être tirée par le secteur civil, et est emblématique de l'inversion des circuits d'innovation traditionnels. Dans ce contexte singulier, les usages de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire doivent impérativement donner lieu à un effort de formation et de programmation. Trois questions semblent s'imposer. La première concerne l'enjeu crucial de formation des armées et de l'ensemble des corps. La cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense annoncée cet été est un mouvement positif, qui permettra de développer une réelle expertise de métier. En parallèle de cette dynamique, comment l'État compte-t-il répondre aux besoins de formation aux nouvelles technologies, induits par l'intelligence artificielle, de l'ensemble de nos forces armées sur le terrain ? deuxième question a trait aux collaborations de recherche comme enjeu de compétitivité. L'objectif est de faire entrer la défense dans les écosystèmes de la recherche publique française, à la fois, par la formation et par la recherche appliquée. Afin de gagner du temps pour développer de meilleures technologies, quelle logique de décloisonnement de la recherche militaire l'État a-t-il prévu afin d'absorber et de collaborer avec les institutions publiques bénéficiant de financements importants en termes d'innovation ? La troisième question porte sur la valorisation croisée des innovations civiles et militaires.

pourront-ils être classifiés facilement, afin de les protéger temporairement ? Enfin, dans quelle mesure ces découvertes de recherche publique pourront-elles bénéficier à nos entreprises françaises ? Ne répétons pas l'erreur commise avec les télécommunications militaires que nous n'avons pas su utiliser dans le domaine civil pour développer la 5 G ! La parole ! La parole est à M. le secrétaire d'État. Il va de soi que, s'agissant d'une technologie aussi importante pour l'industrie et la souveraineté que l'intelligence artificielle, les applications de défense font partie des applications prioritaires.

le Next 40, c'est-à-dire les 40 pépites technologiques françaises dont on espère qu'elles pourraient devenir des licornes. Je ne crois pas qu'une seule d'entre elles ait été financée par le ministère de la défense.

comportements parfois proches de la bestialité qui érodent le lien social et affectif entre les individus. Elle nous conduit à questionner notre rapport éthique à l'intelligence artificielle et à réfléchir à l'utilisation qui en est faite. Implicitement, elle souligne que l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise en soi ; c'est bien son usage qui détermine sa légitimité, ainsi que son apport au bien public. Récemment, un mécanisme de reconnaissance faciale sur la voie publique a été expérimenté pour la première fois en France. De même, une région a manifesté son souhait de tester la reconnaissance faciale par biométrie à l'entrée de lycées. Il est à prévoir que la volonté des collectivités territoriales d'expérimenter ces nouvelles technologies, par-delà la reconnaissance faciale, va probablement s'intensifier à l'avenir. Naturellement, les enjeux d'ordre public pèsent énormément dans leur décision. Pour autant, le recours à des dispositifs fondés sur l'intelligence artificielle ne peut être anarchique. En contrepoint des problématiques sécuritaires se posent des questions majeures en termes tant de respect des droits fondamentaux que de souveraineté numérique. Par conséquent, il est essentiel de fixer démocratiquement une méthodologie et un cadre à l'emploi de ces technologies par la puissance publique. C'est précisément ce cadre qui déterminera leur degré d'acceptation par la population. D'un point de vue juridique, à l'inverse des caméras fixes ou des caméras-piétons, un flou certain demeure sur les usages et les finalités qui peuvent être poursuivis par la reconnaissance faciale et les technologies à venir. Une réflexion sur une éventuelle modification législative et réglementaire paraît, pour le moins, s'imposer. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, mon interrogation est assez simple : entendez-vous ouvrir un véritable débat public sur l'utilisation de la reconnaissance faciale et, plus globalement, sur l'ensemble des technologies futures ayant un impact sur la vie privée, auxquelles pourraient d'ailleurs recourir les collectivités ? Par ailleurs, envisagez-vous de mieux encadrer juridiquement leur usage ? L'équilibre à trouver entre impératif sécuritaire, libertés individuelles et utilisation éthique de l'intelligence artificielle est particulièrement subtil et important

sûrement pas le plus probable, consiste en un déploiement de l'intelligence artificielle aboutissant à la destruction massive d'emplois. Selon un deuxième scénario, peut-être plus sournois, l'intelligence artificielle serait capable de réaliser des tâches de plus en plus complexes, et de s'adapter et d'analyser plus vite que nous ; les emplois peu ou faiblement qualifiés, voire les emplois intermédiaires, seraient alors massivement touchés. Mes questions sont les suivantes, monsieur le secrétaire d'État. Avez-vous identifié les activités et les métiers les plus menacés par le déploiement de l'intelligence artificielle ? Quelle est la stratégie du Gouvernement à Quel accompagnement proposer aux employés peu qualifiés des secteurs de services, qui vont devoir monter en gamme ? Quelles actions envisagez-vous pour diffuser une culture de l'adaptabilité au travail, en France ?

certains métiers fortement répétitifs- vous avez parlé de la banque, on peut aussi penser à la distribution ou à certains secteurs industriels -sont effectivement menacés par l'intelligence artificielle, qui traite très bien les tâches répétitives. Cela concerne aussi des métiers plus élevés, dans lesquels il y a beaucoup de données à traiter ; je pense

Ayant organisé ici même, en juin dernier, avec mes collègues Monique Lubin et Olivier Jacquin, un colloque sur la problématique du travail numérique et les risques de formation d'un « cyberprécariat » dépourvu de droits sociaux,

Le récent numéro de l'émission a opportunément confirmé nos craintes sur la destruction de la citoyenneté sociale des travailleurs, chère au regretté Robert Castel. En effet, par leur modèle de développement, les sociétés multinationales que nous connaissons bien- Uber, Amazon, Google, et -prospèrent sur un vide juridique, que votre gouvernement entretient. Ce vide juridique permet à ces entreprises de ne pas payer de cotisations sociales patronales, en faisant croire aux autoentrepreneurs recrutés qu'ils sont indépendants.

Des microtâches sont réalisées en Asie, en Afrique et en Europe- en France même -par ce qu'Antonio Casilli appelle les « travailleurs du clic », des travailleurs du numérique sous-payés et complètement invisibles pour le droit du travail. Et tout cela au service de la machine, de l'intelligence artificielle, qui dévoile ainsi son vrai visage. Il nous faut donc réfléchir à une fiscalité qui permettrait d'imposer les plateformes sur le fondement du travail invisible de ces usagers, et à un dispositif pour rémunérer la fiscalité est aussi une question de souveraineté. Au regard de l'augmentation du tâcheronnage numérique, allez-vous changer de braquet, et imposer à ces entreprises un cadre beaucoup plus strict et protecteur, afin d'enrayer cette évolution inquiétante du travail ?

il y a aussi un gisement d'opportunités ; dans certains quartiers, l'économie ubérisée a créé de l'emploi et a permis à des gens de se rapprocher de l'emploi. De toute évidence, il faut poser un cadre- on ne peut pas être dans le non-droit total -, mais

député Cédric Villani a largement ouvert le débat public et politique, sur l'urgence qu'il y a, en France et en Europe, à amplifier considérablement les moyens et le soutien au développement de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il s'agit, vous l'avez dit, d'un enjeu majeur pour notre indépendance et notre souveraineté futures. Cédric Villani tente de nous convaincre qu'il n'est pas trop tard pour entrer dans le jeu de la compétition mondiale ; j'en accepte l'augure, et je me félicite des moyens, même s'ils restent insuffisants, débloqués par le Président de la République- un milliard et demi d'euros -pour mettre un coup de pression et encourager le développement de l'intelligence artificielle en France et en Europe.

Bien sûr, le rapport a cherché à proposer, avec humilité, est-il précisé, les fondements d'un cadre éthique pour le développement de l'intelligence artificielle et du débat dans la société.

Déjà, des voix s'élèvent pour affirmer que, si nous sommes trop rigides dans notre conception de l'éthique et des valeurs, cela bridera les initiatives des chercheurs, et nous courons alors le risque de prendre un retard concurrentiel, sur le plan technique, par rapport à d'autres pays. Comment définir, selon vous, les bornes de l'acceptable, voire de l'exigence de notre éthique ? Comment trouver, dans un contexte de concurrence scientifique mondialisée, d'une part, le respect de notre éthique et, d'autre part, l'avancée scientifique de pays qui n'ont pas la même interprétation des valeurs que nous ? Ma deuxième question concerne l'accompagnement juridique de l'intelligence artificielle, et tout particulièrement celui de la responsabilité civile et morale des actes provoqués par l'algorithme. Jusqu'où faire confiance à la décision du matériel porteur de ces algorithmes ? N'y a-t-il pas des domaines qui comportent des limites, au-delà desquelles la décision humaine doit reprendre la main ou le relais de la décision ?

C'est un peu le dernier wagon qui part, mais on peut encore monter à bord. Pourquoi suis-je persuadé qu'il n'est pas trop tard ? Parce que nous avons la matière première : les cerveaux.

Sur la question des valeurs, je pense avoir en partie répondu tout à l'heure. Il faut trouver la ligne de crête, être capable de développer nos propres champions sans abandonner nos valeurs. Ce n'est jamais facile et il n'y a pas de règle préconçue qui s'applique. Cela dit, il faut, au minimum, libérer les expérimentations-

C'est avec un oeil de juriste que j'ai décidé d'aborder le débat que nous avons aujourd'hui. Le développement des intelligences artificielles fait partie des plus grandes avancées scientifiques de l'histoire de l'humanité. Cette révolution technologique a de plus en plus d'impact dans nos vies quotidiennes, on l'a vu. Imaginer les applications matérielles des intelligences artificielles peut susciter l'émerveillement, mais il nous faut aussi examiner des cas pratiques.

En tant que législateurs, nous devons nous interroger sur la place que prendront les intelligences artificielles dans notre droit. Qui devrait-on considérer comme pénalement responsable, lors d'un accident grave causé par une voiture autonome ? Le conducteur ? Le propriétaire ? Le constructeur ? L'informaticien ? Ou encore l'auteur des algorithmes ? On considère aujourd'hui que le conducteur doit toujours être en mesure de prendre le contrôle de sa voiture. Il serait donc en théorie responsable en cas d'accident, mais qu'en serait-il si les véhicules devenaient totalement autonomes ? La même question pourrait se poser pour les intelligences artificielles prédictives en matière militaire.

Les militaires ne veulent pas dépendre de l'incontrôlable, ils veulent rester maîtres de toute leur stratégie. La technologie évolue désormais si vite que nous nous

Pour l'avenir, un régime permanent doit être élaboré par ordonnance, dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 12 du projet de loi d'orientation des mobilités. J'ajoute un élément moins technique : la question que vous posez est

Les Gafama sont arrivés dans le domaine de la santé avec une dynamique d'influence et de diffusion de valeurs qui ne sont pas à proprement parler humanistes. Leur avance industrielle peut avoir des conséquences sur les modalités de diffusion de l'intelligence artificielle et

En France, les données de santé sont et resteront protégées, mais des collectes de données se font via des applications ou des objets connectés, et ces données sont transmises à des entreprises privées sans aucun contrôle. D'autre part, des utilisateurs français pourraient à l'avenir demander à importer une solution d'intelligence artificielle élaborée à l'étranger et non autorisée en France. Sachant que ces entreprises ne respecteront pas forcément les règles éthiques en vigueur en France et en Europe, il est évident qu'il faut organiser un contre-pouvoir au développement des Gafama dans le secteur de la santé. Monsieur le secrétaire d'État, comment faire en sorte que les Gafama ne mettent pas la main sur les données de santé des Français ? Quelle stratégie envisagez-vous de mettre en oeuvre pour préserver le système de santé français face aux géants américains ?

Mme Florence Lassarade, pour la réplique. L'exploitation des données et leur protection sont un sujet très important. Sur le marché noir du net, les données médicales frauduleusement acquises peuvent se monnayer vingt fois plus cher que les données bancaires Merci, Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour conclure ce débat passionnant sur les enjeux politiques, économiques, mais aussi éthiques, de l'intelligence artificielle, je souhaite revenir sur les principaux points que nos échanges ont évoqués. Je me félicite tout d'abord de l'intérêt suscité par ce sujet d'actualité, proposé par le groupe RDSE, qui concerne tous les acteurs et tous les territoires. En introduction, mon collègue Yvon Collin, instigateur de ce débat, a bien insisté sur le développement spectaculaire des technologies d'intelligence artificielle dans le monde actuel. Il a souligné en particulier la place prépondérante des États-Unis et de la Chine, et- hélas ! -le retard européen en la matière. Vous l'avez également souligné, monsieur le secrétaire d'État, nous vivons aujourd'hui à l'époque des algorithmes et des machines apprenantes. Si l'intelligence artificielle a été inventée au tournant de la Seconde Guerre mondiale, les changements se sont vraiment accélérés depuis vingt ans, à un rythme exponentiel, au point de donner parfois le vertige. Cette révolution technologique tend à renforcer le clivage entre des zones urbaines hyperconnectées, qui ambitionnent de devenir des « villes intelligentes », et des territoires, souvent ruraux, qui, pour des raisons géographiques, économiques ou démographiques, restent en marge de cette transformation. Pourtant, les territoires ruraux peuvent tirer un grand parti des applications de l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la santé, ces technologies peuvent ainsi contribuer à faire des prédiagnostics à partir des données médicales des patients ou dans le cadre de consultations à distance, alors que la pénurie de médecins généralistes ne pourra être résolue que dans plusieurs années. Les façons de travailler sont également en plein bouleversement, avec avec des conséquences qui pourraient profiter à des territoires éloignés des grands centres urbains et de tous les inconvénients qu'ils entraînent- surdensité, saturation des réseaux de transport, stress, pollution, voire troubles à l'ordre public ... Nous touchons là à une question structurante de l'aménagement du territoire de demain, un sujet cher à notre groupe. Le rapport Villani, cité plusieurs fois, contient des développements très intéressants sur l'agriculture augmentée, domaine dans lequel la France pourrait devenir un leader. À l'heure du changement climatique et de la remise en cause de notre modèle agricole, l'agriculture a grandement besoin de technologies de big data pour rester productive, tout en tenant compte des impératifs de protection de l'environnement et de la biodiversité. Par exemple, un meilleur suivi des rendements ou des troupeaux permettra d'améliorer le bilan énergétique et d'optimiser l'utilisation d'intrants. L'intelligence artificielle pourrait même contribuer à faire émerger de nouveaux modèles de valeur et à améliorer le dialogue entre les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire. Ce potentiel d'innovation ne doit pas faire oublier les aspects plus préoccupants du développement de l'intelligence artificielle. Le livre récent du philosophe Gaspard Koenig,, Gaspard Koenig,, montre les risques de dépossession et de déresponsabilisation des individus lorsque nos vies seront entièrement façonnées par l'intelligence artificielle, ou encore les opportunités, mais aussi les dangers, liés à la police et à la justice prédictives.

En revanche, l'Europe doit mobiliser beaucoup plus de moyens pour combler son retard technologique. Le 11 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé un financement de 50 millions d'euros pour créer un réseau européen de recherche en intelligence artificielle, dans le cadre du programme Horizon 2020. C'est bien trop peu ! Monsieur le secrétaire d'État, vous avez évoqué la nécessité de constituer de solides équipes de recherche et de pouvoir les conserver en Europe. Dans des secteurs comme l'énergie, la santé ou les transports, nous disposons du savoir-faire de la taille critique pour faire émerger des champions européens. Je salue également les initiatives comme le projet de supercalculateur ou encore l'agence européenne pour l'innovation de rupture. Vous avez mentionné la politique commerciale de l'Union européenne. On pourrait également penser à sa politique de concurrence, dont était chargée la commissaire Margrethe Vestager, qui empêche parfois de faire émerger des champions continentaux. Nous devons progresser sur ce point, afin de pouvoir réaliser « l'Airbus de l'intelligence artificielle car nous ne pouvons nous résigner à laisser l'Europe à la traîne, s'agissant d'une question aussi fondamentale pour notre économie et pour notre souveraineté. Permettez-moi de conclure mon propos avec une citation du cinéaste et humoriste américain, Woody Allen, lequel « l'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine » ...